ma collègue Olivia Richard et moi même avons été enregistrées comme ne prenant pas part au vote, alors que nous souhaitions voter pour. Par ailleurs, lors des scrutins publics n° 48 et n° 54, sur des amendements tendant à supprimer respectivement les articles 6 et 7 du PLFSS pour 2025, ma collègue Christine Herzog a été enregistrée comme votant contre, alors qu’elle souhaitait voter pour. Je vous remercie

de sécuriser les six taxes sur les installations nucléaires de base, dans le contexte du regroupement de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), d’une part, et de l’avancement de la procédure d’autorisation de création,

prévue pour le 1 janvier 2025 alors même que de nombreux salariés en réclament le report. Le comité social et économique (CSE) de l’IRSN et son intersyndicale ont ainsi demandé, le 12 septembre dernier, un report d’un an de cette fusion, déplorant un délai trop court pour son entrée en vigueur à la date prévue. Ils ont notamment fait valoir que le projet d’organisation transitoire proposé avait été élaboré à la hâte au regard de la date de mise en œuvre. Le CSE de l’IRSN a également alerté le collège de l’ASN « sur des constats inquiétants d’une absence de maîtrise et d’une certaine improvisation dans la conduite du projet

Des incertitudes subsistent aussi sur le devenir des activités de recherche conduites par l’IRSN au sein de la nouvelle entité. Pire encore, le rapport général de la commission des finances souligne que le Gouvernement évalue les conséquences de cet article à un gain de 60 millions d’euros pour l’État ; une perte équivalente pour les autres administrations publiques découle directement de la fin de l’affectation de la contribution de radioprotection et de sûreté nucléaire à l’IRSN. C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement de suppression

En effet, les installations nucléaires ne commencent leur activité qu’après la publication de leur autorisation de mise en service, délivrée par l’Autorité de sûreté nucléaire. Avant la mise en service, elles sont en construction, n’accueillent pas de matières nucléaires et ne produisent pas d’énergie. Considérer qu’elles sont déjà en activité est donc inexact, tant scientifiquement que techniquement. Taxer les exploitants alors même que leur installation n’est pas fonctionnelle et ne peut donc générer de chiffre d’affaires est une mesure extrêmement lourde financièrement et entre en contradiction avec la réalité industrielle.

ci n’est pas basée sur le début de l’activité de l’installation, mais sur la publication d’autorisation de sa création, ce qui laisse un délai pendant lequel le constructeur de SMR doit

à l’article L. 542 11 du code de l’environnement. La stabilité dans le temps des ressources de ces GIP conditionne leur capacité à participer

du futur centre de stockage de déchets radioactifs à vie longue Cigéo, a vocation à être temporaire. Il doit logiquement s’éteindre lorsque Cigéo ne sera plus un projet, mais une installation en fonctionnement.

ce texte, « le coût total prévisionnel estimé à environ 2,5 milliards d’euros inclut ainsi 20 % de TVA, soit une charge supplémentaire par rapport au mécanisme actuel de l’ordre de 500 millions d’euros ». Ma question est simple, monsieur le ministre :

de la convergence, ces amendements, de M. Gay et de notre collègue du Rassemblement national.

Avant la crise énergétique, l’accise sur l’électricité était fixée à 32 euros par mégawattheure. Cependant, face à l’envolée spectaculaire des prix de l’énergie, le Gouvernement a choisi de réduire temporairement cette taxe à son minimum légal.

significativement les 32 euros par mégawattheure d’avant la crise, inflation incluse. Une telle perspective est pour le moins inquiétante ; elle est même, à mon sens, illégitime. En effet, cette stratégie reviendrait à faire porter sur l’ensemble des Français le poids de mesures fiscales antérieures qui ont principalement bénéficié à une minorité. En effet, il faut bien rattraper les recettes perdues du fait de la suppression de la taxe d’habitation pour les 20 % des ménages les plus aisés, ou encore la réduction des impôts de production. L’article 7, 7, dans sa rédaction actuelle, s’inscrit dans cette logique. Il accentue les inégalités sociales en faisant peser l’effort de redressement budgétaire principalement sur ceux qui en ont le moins les moyens.

mois de février dernier, alors que les premières alertes budgétaires avaient été lancées, Bruno Le Maire a décidé de revenir sur le principal dispositif du bouclier tarifaire sur l’énergie.

à utiliser une énergie décarbonée, quand, dans le même temps, l’État ne cesse de modifier les règles et de surenchérir les coûts ? L’électricité est désormais l’énergie la plus taxée en France ; elle est devenue une vache à lait pour les finances publiques. La facture d’électricité n’est plus qu’un empilement de taxes, d’accises, de fiscalités en tout genre. Nous l’avons compris, cette mesure n’a que des avantages aux yeux du Gouvernement. En effet, comme pour la TVA, elle rapporte beaucoup et immédiatement.

d’alourdir encore une fois les impôts des Français. Vous soutenez un système profondément déséquilibré, qui nuit à notre économie et alourdit les charges des ménages et des entreprises. Il convient donc de supprimer cet article.

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

faut que l’effort profite d’abord à ceux qui participent effectivement à la transition énergétique et au verdissement du gaz. Quel

aux fournisseurs, qui auront le temps d’adapter leur système facturier aux évolutions décidées dans les différentes lois de finances.

inégalitaires qui soient : elle est acquittée par l’ensemble des ménages, indépendamment de leurs revenus, et pèse donc plus particulièrement sur les travailleurs et sur les foyers les plus précaires. Nous pensons au contraire que l’énergie abonnement et consommation – est un bien de première nécessité. À l’instar d’autres secteurs ou catégories de produits, il est donc impératif qu’elle bénéficie d’une TVA plus avantageuse, ce que permet d’ailleurs la législation européenne. Vous faites le choix de l’austérité ; ne vous cachez pas derrière les textes européens ! L’amendement

seront taxés à taux plein. Ce sont donc les habitants des zones rurales qui seront les plus pénalisés par cette hausse. La fiscalité écologique doit être incitative. C’est pourquoi elle repose sur la consommation – molécules et électrons – et non sur les abonnements. Avec cette réforme, les consommateurs seront taxés à taux plein avant même d’avoir consommé ; les ménages précaires et les ménages sobres seront proportionnellement les

comme le projet de loi de finances le prévoit, un financement pérenne de la péréquation territoriale entre le territoire continental et les zones non interconnectées, tout en sécurisant la compensation intégrale des charges de service public supportées par les opérateurs concernés.

l’article 7, celui ci permet de sécuriser la péréquation territoriale, qui souffre d’un déséquilibre croissant entre les coûts de production dans les ZNI et leur financement actuel, qui repose largement sur le budget général de l’État. L’option retenue par le Gouvernement consiste à mettre en œuvre de nouvelles modalités de compensation des charges de service public en ZNI. en ZNI. La péréquation territoriale avec les ZNI serait sortie du régime standard de compensation intégrale des charges de service public de l’électricité. Elle reposerait désormais sur l’affectation d’une part du produit de l’accise sur les énergies.

de garantir un financement durable de la péréquation territoriale entre le territoire continental et les zones non interconnectées, tout en sécurisant la compensation intégrale des charges de service public supportées par les opérateurs

Cet amendement vise à consolider le financement des opérations liées à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées, en reprenant d’ailleurs une terminologie déjà utilisée en matière de charges de service public.

Monsieur Savoldelli,

Le scrutin est clos.

dans les zones rurales, en remettant en cause le financement des travaux que réalisent aujourd’hui les syndicats d’énergies de France sur 75 % de notre territoire pour assurer la modernisation et la résilience des réseaux. dit on, serait une réponse à un risque juridique lié au droit européen. Pourtant, il n’en est nullement fait état dans l’évaluation préalable des articles du PLF pour 2025, qui ne mentionne qu’un objectif de simplification du droit fiscal en Ce risque juridique est au demeurant infondé, puisque la contribution actuelle versée par les gestionnaires du réseau de distribution (GRD) d’électricité au CAS Facé et l’accise sur l’électricité ne reposent pas du tout sur la même assiette d’imposition, contrairement à ce que j’ai entendu affirmer. Cette réforme entre, de surcroît, en contradiction avec le principe selon lequel tout service public, industriel ou commercial, est financé non par une taxe,

Les comptes d’affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées. » Je soutiens la position de Mme Saint Pé : il existe,

de la réforme du financement du CAS Facé, je soulignerai que le prélèvement d’une fraction de l’accise sur l’électricité de manière uniforme sur l’ensemble du territoire va conduire, malheureusement, à supprimer un dispositif de péréquation et de solidarité territoriale ô combien nécessaire

ne bénéficieront malheureusement plus des mêmes garanties que ceux qui sont situés en zone urbaine. Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cette réforme, d’autant qu’elle n’a fait l’objet d’aucune véritable concertation ni d’aucune étude d’impact préalable. La parole

qu’est ce qui nous assurera que ces fonds seront bien affectés à l’électrification rurale ? Ce qui change, c’est l’origine des financements, puisque les gestionnaires de réseau ne vont plus financer ce fonds, comme ils le faisaient

L. 312 1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité, déterminée sur la base d’un tarif de 1,30 euro par mégawattheure majoré chaque année de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en référence à l’année 2025.

n’ont pas encore reçu l’arrêté de notification du montant qui doit leur être alloué en 2024, en raison d’une difficulté d’interprétation par les services de l’État des dispositions de l’article L.

Michel Canévet, pour explication de vote.

L’objectif, le cap, le solde, les moyens pour y parvenir, cela fait deux mois que je les répète, et encore ici hier, lors de la discussion générale.

d’ester méthylique d’acide gras est, depuis 2022, obligatoire pour toute nouvelle chaudière de type fioul installée, conformément aux dispositions du décret n° 2022 8.

Je rappelle que le fioul est particulièrement utilisé dans des zones où les températures hivernales sont basses, où les réseaux de gaz n’existent pas et où la substitution par une pompe à chaleur C’est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, équipant près de 3 millions de logements, des maisons individuelles pour la plupart. Le développement du biofioul permettrait ainsi de préserver le mode de chauffage des territoires ruraux les plus éloignés, tout en progressant dans la décarbonation.

la facture d’électricité des ménages est devenue disproportionnée par rapport à leurs revenus et l’État a dû mettre en place un bouclier tarifaire pour limiter la hausse. D’autre part, les projets d’énergie renouvelable et de récupération, notamment ceux qui concernent les réseaux de chaleur, ont exercé un attrait sans précédent

et de récupération produites localement et un temps de retour acceptable pour les travaux de rénovation globale, et, d’autre part, au dessous d’un prix plafond qui reste soutenable socialement.

Par cet amendement vous est communiqué le tableau dit de simplification – c’était encore plus complexe avant – concernant les tarifs d’accise sur l’électricité

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, En France, les fabricants de chips, y compris ceux qui produisent des chips artisanales, sont assujettis à l’accise sur les gaz naturels et, contrairement aux autres fabricants de légumes déshydratés implantés dans l’Hexagone, ils ne bénéficient pas du tarif réduit prévu par le code des impositions sur les biens et services. Ainsi, ils restent soumis au tarif normal, tandis que leurs concurrents internationaux, implantés en Belgique, par exemple, supportent une taxation équivalente au tarif réduit français, ce qui leur permet de produire à un coût inférieur à celui de nos fabricants.

Pour cela, il est indispensable d’étendre ce tarif réduit aux fabricants de chips implantés en France, qui sont actuellement les seuls exclus du dispositif. Cette mesure, qui serait peu coûteuse pour nos finances publiques, irait dans le sens de la reconquête du marché français, à l’instar de ce qui se passe dans le secteur de la frite : des usines rouvrent en France depuis que notre fiscalité s’est alignée sur celle de la Belgique. L’amendement

Malgré des charges d’exploitation élevées, sa rentabilité économique est plus élevée de cinq points – 10,4 % contre 5,5 % –, que celle du secteur des transports

et 2022. Ce rapport montre que la détaxe sur le carburant a représenté 203 millions d’euros en 2021, soit 63 % du montant total des subventions publiques accordées à ce secteur. Près de 47 % des subventions au carburant ont bénéficié à des navires de plus de vingt Ces navires industriels captent donc près de la moitié des subventions au carburant de la flotte de pêche française, alors qu’ils ont un impact massif sur les écosystèmes marins et le climat. Ils accaparent les quotas au détriment des pêcheurs artisans et côtiers. Ils sont pourtant deux à trois fois moins rentables que les petits navires pratiquant la pêche aux arts dormants. Dans une optique de transition sociale et écologique du secteur de la pêche, il convient de cesser de subventionner ces navires industriels pour soutenir le développement d’une pêche artisanale sur nos littoraux. cet amendement, nous proposons donc de supprimer en trois ans, par tranches de 30 % les deux premières années et de 40 % la troisième année, le tarif réduit qui s’applique aux produits taxables utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation maritime ou destinés à l’avitaillement d’un navire professionnel. Cette suppression ne concernera ni les entreprises de pêche artisanale exploitant des navires de moins de vingt quatre mètres ni les autorités publiques, qui continueront de bénéficier du tarif réduit en raison de leur rôle spécifique et des contraintes particulières auxquelles elles sont soumises.

une augmentation des objectifs d’incorporation de biocarburants, mais impose aussi l’abandon du double comptage pour les carburants dits de deuxième génération. Il supprime aussi la possibilité d’échapper à ces objectifs une taxe exonératoire, en la remplaçant par une amende

Néanmoins, en limitant la comptabilisation des quantités d’hydrogène délivrées aux véhicules équipés de piles à combustible, le mécanisme exclut une part importante de véhicules qui pourraient constituer des moyens supplémentaires d’engager rapidement cette transformation vers l’objectif de zéro émission

le potentiel industriel de cette filière, on encouragerait le développement de rétrofiteurs et de motoristes nationaux, et l’on soutiendrait les transporteurs aux marges économiques restreintes dans leur décarbonation. Tel est le sens de cet amendement.

monsieur le ministre,

la suppression de cette niche fiscale engendrerait un gain annuel de l’ordre de 700 millions d’euros pour l’État. Ces ressources pourraient être réinvesties dans des solutions énergétiques réellement durables et alignées sur nos ambitions climatiques. En soutenant une mesure de cette ampleur, nous enverrions un signal fort : les politiques fiscales doivent être cohérentes avec nos engagements écologiques et sociaux et cesser de privilégier des pratiques, notamment agricoles, qui aggravent la crise environnementale.

et bas carbone. L’objectif est d’encourager le développement de ces gaz verts, qui sont notamment produits par la méthanisation agricole, le traitement des boues des stations d’épuration ou la valorisation des biodéchets. Ces énergies renouvelables nous permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre,

cette disposition a été supprimée dans la loi de finances pour 2021 : demande de retrait

de verdissement de leurs bâtiments : couverture des parkings extérieurs d’ombrières photovoltaïques ; intégration soit d’un procédé de production d’énergies renouvelables, soit d’un système de végétalisation sur les bâtiments nouveaux ; pose d’ombrières photovoltaïques ou de systèmes de végétalisation sur les bâtiments anciens ; réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires de plus de 1 000 mètres

plus de 100 kilomètres par jour travaillé en moyenne dans le cadre de leur activité professionnelle, selon les mêmes modalités que celles prévues pour les entreprises de transports routiers de marchandises et les exploitants de transports publics de voyageurs. Les difficultés d’accès aux professionnels services de santé sont une préoccupation majeure pour une grande partie de nos concitoyens : selon une récente enquête d’opinion, 80 % d’entre eux s’en inquiètent, en particulier dans les zones rurales. Aussi, pour résoudre ce problème, il est essentiel de soutenir la mobilité des professionnels de santé.